Je regrette que la conférence des présidents n'ait pas accordé d'explications de vote sur un texte aussi important, qui engage notre diplomatie.

C'est la preuve que les textes qui sont examinés, débattus et votés par le Parlement font écho à la vie de nos concitoyens, qui, vous en conviendrez, est malheureusement bouleversée Le Gouvernement a fait des choix clairs et ambitieux : protéger nos concitoyens face au virus, soutenir l'hôpital public et les soignants, faire avancer la société en consacrant des droits nouveaux, réarmer notre protection sociale et organiser la prévention et la protection face à un risque croissant, celui de la perte d'autonomie. Alors que nous arrivons au terme de l'examen de ce PLFSS, avec le dépôt d'une question préalable, qui sera vraisemblablement adoptée dans les prochaines minutes,

a été rehaussé de 3,2 milliards d'euros supplémentaires au cours de l'examen du texte, pour tenir compte des surcoûts liés à la crise du covid et pour accélérer le calendrier de revalorisation salariale de nos soignants. La promesse du Président de la République de répondre à la situation « quoi qu'il en coûte » n'était donc pas une formule ; nous sommes bien au rendez-vous. Par ailleurs, un accord a pu être trouvé entre les deux chambres, sur plusieurs articles, et non des moindres je me satisfais du vote conforme s'agissant du financement de la prime covid pour les salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), ainsi que des revalorisations dans les Cette revalorisation prévoit 183 euros nets de plus par mois au sein des établissements de santé, Ehpad publics et privés non lucratifs, et de 160 euros nets de plus par mois pour le secteur privé lucratif. Quand nous connaissons l'enjeu que représentent le grand âge et l'autonomie dans notre pays, quand nous connaissons l'engagement de celles et ceux qui sont auprès de nos aînés, il ne se trouvera personne sur ces travées pour estimer que cette augmentation de salaire serait injustifiée. Nous pouvons aussi nous féliciter de l'adoption conforme de l'allongement du congé paternité, voté à la quasi-unanimité dans les deux assemblées. Au-delà de ces premiers sujets, un vote conforme a d'ores et déjà été obtenu pour une cinquantaine d'articles. Je pense notamment à la création d'une mission d'intérêt général pour lutter contre les violences faites aux femmes, ou encore à la garantie du tiers payant et du secret pour les frais liés à l'interruption volontaire de grossesse En nouvelle lecture à l'Assemblée, le rapporteur général et le Gouvernement ont apporté des aménagements sur quelques dispositions pour lesquelles un accord avec la Haute Assemblée était tout proche. Je pense, par exemple, à certaines dispositions relatives à la lutte contre les fraudes. L'Assemblée est en revanche revenue, avec l'assentiment du Gouvernement, sur d'autres dispositions que vous aviez votées lors de l'examen de ce projet en première lecture. Je pense ici à l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. De la même manière, s'agissant du financement inédit d'un effort de revalorisation des métiers du domicile, si vitaux pour l'accompagnement des personnes âgées, il nous est apparu indispensable de revenir à un dispositif qui respecte la compétence des départements. Évidemment, nous visons une hausse des salaires sur tout le territoire national ; tel est l'objectif de la démarche que j'ai entreprise. Cependant, ce n'est pas en déresponsabilisant les conseils départementaux que nous aurons une meilleure politique de l'autonomie. Je veux d'ailleurs réaffirmer clairement, car je sais à quel point vous y êtes attachés, que l'objet de cette aide est bien de financer l'augmentation salariale, sans ambiguïté. En agréant l'avenant 44 à la convention

quelle que soit leur affiliation à un régime de sécurité sociale : les salariés et les non-salariés agricoles sont donc couverts, sans ambiguïté. Voilà qui ne remet aucunement en cause le rôle fondamental de la MSA dans les territoires, en faveur de la mise en oeuvre des politiques de santé, de prévention et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. La création de la branche autonomie ne dépossède en rien les caisses de la MSA de leurs missions et de leurs actions en soutien à la perte d'autonomie. Enfin, le rétablissement des dispositions relatives à la reprise des dettes d'hôpitaux permettra d'apporter 13 milliards d'euros de soutien à notre système de santé. Mesdames, messieurs les sénateurs, les débats ont parfois été vifs, toujours passionnés, mais il faut nous réjouir de voir que l'hôpital public, les soignants, la famille, le grand âge et l'autonomie mobilisent pleinement les représentants de la Nation. Ces débats ne s'achèvent pas, bien sûr, avec ce PLFSS ; le projet de loi sur le grand âge et l'autonomie permettra de continuer à faire avancer, au-delà de la crise que nous traversons, le renforcement de la protection sociale de nos concitoyens tout au long de la vie. La parole

sont particulièrement contraints. Je limiterai donc mon propos à l'essentiel. Tout d'abord, madame la ministre, comme votre collègue Olivier Dussopt nous l'avait annoncé lors de la première lecture, le Gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale des amendements

de la dégradation des hypothèses macroéconomiques. La prévision de croissance du PIB pour 2021 ne serait que de 6 %, contre 8 % prévus auparavant. De même, la croissance de la masse salariale

Quelques-unes de nos initiatives ont été conservées par l'Assemblée nationale à l'occasion de la nouvelle lecture. Je pense, par exemple, à la mise en place de la branche autonomie, comme Mme la ministre l'a Ont été maintenues les précisions apportées au rôle de la CNSA en matière de soutien à l'habitat inclusif, les conséquences qu'implique la création d'une nouvelle branche pour la caisse centrale de la MSA, dans une rédaction un peu remaniée par le Gouvernement, le Gouvernement, et surtout le principe d'une conférence des financeurs du soutien à l'autonomie chargée de formuler des recommandations sur le financement des mesures nouvelles les députés ont toutefois aligné son périmètre sur celui du conseil de la CNSA, ce qui est peut-être regrettable ; nous pensions pouvoir l'élargir un peu. Je pense aussi à plusieurs dispositifs anti-fraude introduits au Sénat : l'annulation automatique des obtenus de manière frauduleuse, mesure sur l'initiative de Mme Goulet ; l'extension à cinq ans de la prescription des indus frauduleux de la sécurité sociale, sur l'initiative de la commission ; l'instauration d'une dérogation au délai maximal de sept jours pour le paiement par l'assurance maladie de professionnels de santé convaincus de fraude à des fins de contrôle, sur l'initiative de la commission ; ou encore le déconventionnement d'office en cas de récidive en matière de fraude par un professionnel de santé, toujours

que nous nous retrouverions certainement fin 2020 pour prolonger ce dispositif. Nous y sommes ! Ce dispositif sera sans doute de nouveau prolongé fin 2022, car il répond à l'équilibre économique des filières concernées. Il serait donc beaucoup plus raisonnable de pérenniser l'exonération TO-DE, afin de donner une véritable visibilité aux filières concernées, plutôt que de leur donner l'impression d'un sursis permanent. Au-delà de ces sujets sectoriels, nos différends avec l'Assemblée nationale portent aussi sur des questions fondamentales pour l'équilibre des finances sociales. Je pense à la compensation à la sécurité sociale de l'ensemble des pertes de recettes de ces deux dernières années, en application des principes définis dans le rapport dit « Charpy-Dubertret » sur la rénovation des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. Je pense aussi à la révision pour 2020 de la compensation de l'État au titre de la prise en charge de l'Agence nationale de santé publique (ANSP), dite Santé publique France, dont le budget est passé en un an de 150 millions d'euros à 4,8 milliards

En somme, le désaccord reste entier pour l'ensemble des différends qui ont abouti à l'échec de la commission mixte paritaire. Or, comme vous le savez, il s'agit de sujets qui posent de sérieux problèmes de principe. Ainsi, comment imaginer revenir à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale si on la leste de charges qui ne sont pas les siennes, comme celles de Santé publique France, si on multiplie les entorses à la loi Veil et si on se refuse à engager la concertation sur des réformes qui seront, et sont déjà nécessaires ? ? Comment éteindre un jour la dette sociale si l'on commence à faire financer n'importe quoi par la Cades ? Avec un tel précédent, il ne faut pas s'étonner d'entendre déjà certains ministres-

la commission a considéré qu'il était préférable d'acter la fin du dialogue utile entre les deux assemblées. C'est pourquoi elle proposera au Sénat d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable. Bravo ! La parole est

Malgré les dépenses liées au covid, ce PLFSS accorde une augmentation de salaire très importante aux soignants en hôpital et en Ehpad, pour 9 milliards d'euros, ainsi que d'autres avancées significatives. Nous regrettons le rejet par l'Assemblée nationale de nombreuses mesures adoptées par le Sénat- comme l'a dit le rapporteur général

Certaines dispositions du Sénat ont été maintenues, notamment les mesures visant à renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude, l'annulation du numéro de sécurité sociale obtenu frauduleusement, l'expérimentation d'une carte biométrique et et le déconventionnement de praticiens fraudeurs. La réunion d'une conférence de financeurs de la politique de soutien à l'autonomie a été conservée. Il s'agit de prévoir les financements supplémentaires de la cinquième branche. Les besoins urgents s'élèvent à 2 milliards d'euros en 2021, 6 milliards en 2024 et 10 milliards en 2030, avec un doublement progressif du nombre de soignants, infirmiers, aides-soignants en Ehpad, tout en améliorant l'attractivité des carrières et la formation. Le renforcement du maintien à domicile est une priorité absolue, nécessitant un grand plan national d'adaptation des logements à la dépendance

de mesures paramétriques et l'accélération de la réforme Touraine. Les circonstances actuelles ne sont pas favorables à l'adoption d'une telle réforme, mais, compte tenu du vieillissement de la population et du déficit très important la branche retraite, qui s'élève à 8 milliards d'euros en 2020 et davantage en 2021, des mesures seront nécessaires pour maintenir le niveau des retraites. Nous étions favorables à la différenciation du taux de contribution exceptionnelle selon le caractère lucratif ou non des OCAM et à la hausse du taux de contribution en 2021, pour porter la contribution à 1 milliard, au lieu de 500 millions revanche, mon groupe n'était pas opposé à une reprise d'une partie des 13 milliards d'euros de dette hospitalière par la Cades, afin que les hôpitaux retrouvent une capacité d'investissement.

en charge par la Cades aujourd'hui. Il en est de même pour une partie des dépenses exceptionnelles de l'Agence nationale de santé publique. Il nous semble qu'un travail de conciliation aurait pu être réalisé, en particulier en cette période difficile pour le milieu en particulier en cette période difficile pour le milieu hospitalier dans notre pays, notamment sur les 13 milliards d'euros d'investissements attendus. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants s'abstiendra sur la motion de rejet.

avant toute chose, notre groupe tient à saluer les quelques avancées du PLFSS : le Ségur de la santé, l'allongement du congé paternité, les maisons de naissance ou l'avancement du versement de la prime de naissance. Hélas, face à ces quelques pas en avant, en cette fin de navette parlementaire, ce texte maintient sa trajectoire austéritaire. Voici quelques exemples : l'hôpital est toujours sommé de réaliser 800 millions d'économies ; la dette des hôpitaux n'est pas reprise par l'État ; la cinquième branche ne dispose pas de financements nouveaux,

Notre groupe, après avoir fait adopter quelques mesures lors de l'examen au Sénat, regrette que celles-ci aient été supprimées par nos collègues députés. Parmi ces dispositions figuraient des mesures pour lutter contre le non-recours aux prestations sociales- elles ont été supprimées par l'Assemblée -et le refus du transfert de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vers la sécurité sociale, nouveau désengagement de l'État dénoncé par les acteurs de la solidarité- rétabli -, sans parler du rétablissement de la surcotisation salariale des sapeurs-pompiers, alors que sa suppression avait été largement soutenue et votée sur l'ensemble de nos travées. Au-delà de la suppression de nos amendements, nous assistons à un détricotage mécanique et systématique du travail du Sénat exercé par les députés de la majorité présidentielle. Cela fera l'objet de la question préalable. Le groupe écologiste regrette également le rejet d'autres dispositions que nous avions soutenues, comme la compensation à son coût réel de Santé publique France par l'État et le refus de faire porter à la Cades la reprise du tiers de la dette des hôpitaux,

prime covid a créé des disparités et des injustices. Sur les rangs de nos deux assemblées, des amendements ont été déposés pour pallier les inégalités et revaloriser les salaires de tous les oubliés du Ségur de la santé,

et du risque d'une crise inédite, alors que la « digue du domicile » permet à l'hôpital- lui-même sinistré -de tenir en période de pandémie. Non seulement, madame la ministre, votre gouvernement ne tire aucun enseignement de cette crise, mais il contribue même à l'approfondir ! Depuis le premier examen vous venez de prier la branche du domicile de retourner à la table des négociations, alors que, après de nombreux rapports et de longues négociations, les partenaires sociaux, employeurs et syndicats, s'étaient mis d'accord sur une réforme ambitieuse qui posait enfin,

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne regrettera pas, en revanche, que certaines mesures introduites par la majorité sénatoriale, telles que la tentative d'accélérer la contre-réforme des retraites,

La clause de sauvegarde et les mécanismes actuels de soutenabilité des dépenses de médicaments face au développement des biothérapies, à l'article 17, ou encore l'expérimentation de l'ouverture de la pratique des IVG instrumentales par les sages-femmes, à l'article 34 ont ainsi été supprimés lors de l'examen. Il en va de même pour l'article 27 portant sur la reprise partielle de la dette des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Et que dire de l'amendement présenté en fin d'examen du projet de loi et visant à reporter l'âge d'ouverture des droits à la retraite, La conclusion allait de soi : les divergences entre les représentants de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat étaient bien trop profondes pour que la commission mixte paritaire parvienne à trouver un accord. C'est le quatrième PLFSS que je suis, et c'est la quatrième fois qu'il se termine ainsi. Pour autant, et bien que vous scandiez le contraire, les députés, en deuxième lecture, ont su faire le jeu du bicamérisme et accepter certaines de vos propositions. Je pense notamment aux mesures de lutte contre la fraude sociale, comme l'annulation automatique du NIR obtenu frauduleusement, à l'article 43 BB, la dérogation à l'obligation de paiement sous sept jours de l'assurance maladie en cas de fraude, à l'article 43 G, au déconventionnement d'office des professionnels de santé condamnés pour fraude à plusieurs reprises, à l'article 43

Des députés serviles, une administration omnipotente : telles sont, en commission des affaires sociales, les deux raisons qui justifieraient le rejet d'une discussion sur le PLFSS. Dois-je vous rappeler qu'il constitue l'un des exercices les plus singuliers depuis sa création en 1996, tant au vu de la pandémie mondiale qui nous frappe et de son impact sur les finances sociales qu'en raison des transformations structurelles auxquelles il donne une traduction législative concrète ? En désignant des boucs émissaires, vous vous exonérez de l'examen de ce projet de loi en deuxième lecture. Mes chers collègues, j'entends vos oppositions de principe, qui, à force, ressemblent à des postures politiciennes. Mais quelle tristesse d'écorner encore, et pour la énième fois, le bicamérisme Ce texte nous donnait pourtant matière à débattre, et c'est bien là l'essence même de notre fonction. Avec une telle posture, vous assumerez de dire aux Français que les grandes transformations structurelles proposées ici, à l'instar de la traduction du Ségur, avec notamment la revalorisation des salaires, l'augmentation de l'Ondam, l'allongement du congé de paternité, ou encore la création de la cinquième branche ne sont pas la hauteur de vos quelques propositions non retenues à l'Assemblée nationale. Vous l'aurez compris, nous voterons contre cette question préalable.

Pour ceux qui s'y intéressent, le PLFSS est, chaque année, un moment fort du calendrier législatif de notre assemblée. Cette fois, plus que les autres, il marque nos débats par son emprise directe avec la crise sanitaire et économique que nous vivons.

de nos travaux sur ce texte. Pourtant, nous sommes convaincus qu'un consensus pouvait, aurait pu être trouvé avec les députés. Quelques sujets nous rassemblent : pas moins de 42 articles ont été adoptés conformes par les deux assemblées en première lecture.

Sur ce sujet, c'est bien le débat qui nous a permis d'aboutir à un vote conforme à la quasi-unanimité, et ce n'était pas gagné au vu des réticences au sein de notre hémicycle. Pourtant, nous pouvons nous en réjouir, et même en être fiers. La presse titrait déjà sur la résistance des « papys et mamies du Sénat » ... Nous avons montré que, loin de ces caricatures, le Sénat est prêt à accompagner l'évolution d'une société dans laquelle les pères souhaitent prendre toute leur place à côté de leur enfant. Enfin, certaines modifications opérées au Sénat ont été conservées par l'Assemblée nationale. Parmi celles-ci, je note particulièrement : l'allégement des cotisations et contributions sociales pour les employeurs et travailleurs indépendants touchés par la crise ; les dispositions relatives à la pratique sportive en entreprise, auxquelles nous tenions beaucoup nous tenions beaucoup ; et la possibilité pour les maisons de naissance, par exemple, de réaliser des missions de prévention et de constituer des lieux de stages. Néanmoins, force est de constater que de profonds désaccords ont subsisté, et qu'ils n'ont pas permis aux rapporteurs de l'Assemblée et du Sénat d'aboutir à un texte commun lors de la commission mixte paritaire. Les mesures relatives aux retraites ont cristallisé les oppositions. Mon groupe s'est exprimé clairement sur ce sujet lors de la première lecture : ces amendements n'avaient, selon nous, pas leur place dans ce texte. Si cette réforme doit prochainement aboutir, et nous partageons le constat de cette exigence, elle mérite une concertation et un débat approfondis, dans le cadre d'un projet de loi qui lui sera dédié, même si, pour l'instant, cette Sur d'autres points, nous regrettons le rejet par l'Assemblée nationale de propositions que nous jugeons nécessaires et que nous aurions souhaité voir inscrites dans le texte final. Je pense, par exemple, au stock de quatre mois minimum pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Le Gouvernement souhaite deux mois maximum et appelle au réalisme, permettez-moi de rappeler ce qu'est la réalité : 45 % des personnes confrontées à des pénuries de médicaments ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d'y renoncer. ! Ces pénuries ne font que s'aggraver : 3 200 médicaments à intérêt thérapeutique majeur manquaient en 2020, alors qu'ils n'étaient que 40 en 2008 ! Notre rapport sur le sujet, publié voilà déjà deux ans, appelait à des réponses rapides et ambitieuses. Nous persistons donc naturellement dans cette voie. D'autres trop nombreux apports retoqués ont été rappelés par le rapporteur général. Compte tenu des blocages qui persistent et du vote à venir d'une motion de rejet, nous ne pouvons espérer voir émerger un consensus sur ce texte. Victor Hugo disait : « La France gouvernée par une assemblée unique, c'est-à-dire l'océan gouverné par l'ouragan. Le bicamérisme garantit l'existence d'une authentique discussion législative, qui privilégie l'esprit de sagesse et concourt à la qualité de la loi. Attaché à ces valeurs, le groupe RDSE aurait souhaité voir les débats se poursuivre et votera donc contre la motion tendant à opposer la question préalable.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le ministre de la santé, avec qui nous n'avons pas eu l'honneur d'échanger en première comme en seconde lecture de ce PLFSS, a défendu devant nos collègues députés un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qu'il a qualifié d'« exceptionnel », », ajoutant qu'ils auraient pu faire d'autres choix : « Serrer la vis, réduire la voilure ou couper le robinet [ ...] Ce choix de l'austérité, dont les conséquences auraient évidemment été dramatiques, nous ne l'avons pas fait. Qui est dupe de ce recours à l'auto-persuasion ? Certainement pas les personnels hospitaliers ni ceux du secteur médico-social ! L'Ondam fixé pour 2021 suit la même logique que tous ceux qui ont été votés depuis 2008, à savoir une progression, à hauteur de 2,4 %, inférieure à l'évolution tendancielle des dépenses de santé, provoquant, une fois de trop, des coupes budgétaires terribles pour notre système de santé. Cette fois, ce sont 4 milliards d'euros qui sont rognés, dont 800 millions pour l'hôpital. Moi, madame la ministre, j'appelle cela une cure d'austérité Le langage de vérité est de dire que vous continuez à considérer l'hôpital comme une variable d'ajustement de votre politique de restrictions budgétaires. Comment construire le PLFSS 2021 sans prendre en compte les réalités de terrain ? Entre 2008 et 2017, 10 % des établissements ont été fermés 15 % des lits ont été supprimés. Et vous continuez dans cette funeste logique. Bien que la pandémie ait mis en évidence un manque de lits criant, et pas seulement de lits de réanimation, 13 établissements de santé viennent encore de perdre des places. Votre machine à restructurer l'offre hospitalière ne s'arrête pas là. Ainsi, à Marseille, le centre hospitalo-universitaire de Sainte-Marguerite doit faire face au démantèlement programmé de sa pharmacie, après la fermeture des urgences et la disparition du service de réanimation. En Île-de-France, la réduction des capacités hospitalières se poursuit avec la construction de l'hôpital Nord, qui se traduira par la fermeture des hôpitaux Bichat et Beaujon. À la clé, la disparition de 300 à 400 lits Alors que la covid-19 a démontré combien il fallait repenser la place de nos aînés en situation de dépendance dans nos structures d'accueil et de soins, le plan Gériatrie est toujours d'actualité à l'AP-HP avec la fermeture de 40 % des lits de soins de longue durée ! Ces exemples, parmi des centaines d'autres, sont la traduction directe, madame la ministre, des PLFSS successifs, dont celui de 2021. Ce projet de loi de financement n'a décidément rien d'exceptionnel. Vous avez annoncé vouloir améliorer l'attractivité des métiers à l'hôpital, mais les étudiantes et les étudiants en santé, les soignants, les médecins n'en peuvent plus et démissionnent sans bruit, à cause des conditions de travail dégradées par des décennies de réduction des budgets. Vous avez annoncé vouloir revaloriser les salaires de celles et ceux qui ont été en première ligne. Pourtant, 50 000 agents du secteur médico-social, dont le secteur de la psychiatrie, sont exclus de la revalorisation salariale du Ségur de la santé. Ces hommes et ces femmes se mobilisent pour faire entendre cette injustice. Nous demandons qu'ils soient enfin entendus. Alors que, depuis de nombreux mois, la branche de l'aide, de l'accompagnement et des soins à domicile était en négociation sur la classification et les rémunérations, et malgré l'unanimité entre les organisations syndicales de salariés et la représentation des employeurs, l'avenant 43- je parle bien du 43 -, qui prévoit un rattrapage et une augmentation de salaire n'a pas reçu l'avis favorable du Gouvernement, car considéré comme trop onéreux. Le « quoi qu'il en coûte » ne s'applique décidément pas à tout le monde Pour ce 75 anniversaire de la sécurité sociale, nous espérions que l'État, conformément à ses engagements, compense à l'euro près les pertes de recettes et les nouvelles dépenses infligées à notre système de protection sociale. Malheureusement, il n'en est rien. Nous avions déposé de nombreux amendements en première lecture. Très peu ont été adoptés, pour être directement rejetés par l'Assemblée Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera donc contre ce budget de la sécurité sociale pour 2021, largement déconnecté des besoins sociaux, et qui continue à affaiblir notre système de protection sociale de haut niveau, tournant le dos, chaque jour davantage, à une société solidaire. La parole

avec un projet qui est marqué essentiellement par votre méthode parlementaire ; je vous le dis directement : elle nous pose problème

de son premier examen, et encore lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes allés beaucoup plus loin. Vous avez écarté et balayé de nombreux ajouts du Sénat, qui n'étaient pas d'un fait majoritaire évident dans cette assemblée, mais qui avaient été adoptés largement parce qu'ils apportaient une construction réfléchie, utile, parlementaire à la qualité du texte. C'est cela que nous dénonçons, madame la ministre,

montre que vous imposez la seule volonté de l'exécutif. Si c'était un parlementaire ou simplement un groupe parlementaire de l'opposition qui le dénonce, vous diriez que c'est le jeu démocratique, sauf que ce constat, vous le savez, est largement partagé au sein du groupe du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est un constat que vos députés font également en partie ; c'est le constat, je vous le dis très tranquillement, d'une démocratie parlementaire que, malheureusement, vous altérez. altérez. Dans ces conditions, nous comprenons la question préalable qu'a déposée le rapporteur général de la commission, même si nous, par principe, nous préférons poursuivre le débat. Vous le voyez, nous ne désespérons jamais. je voudrais soulever quelques points seulement qui illustrent, dirai-je, la profondeur du désaccord. Sur la question des compensations, le rapporteur l'a très bien dit,

de l'État : le budget social devient une annexe du budget de l'État et vous transférez sur le système de protection sociale les déficits qui sont ceux de l'État.

du financement de l'Agence nationale de santé publique à l'assurance maladie. Vous avez dit à l'Assemblée nationale que c'était pertinent, compte tenu de la nature des activités de l'Agence. Mais non ! Mais non ! Les faits sont têtus : les prérogatives de l'Agence nationale de santé publique sont en large partie des prérogatives d'État- la veille et la sécurité sanitaires, par exemple -, et non pas des prérogatives de l'assurance maladie. J'y insiste, il est très difficile de débattre quand la réalité des faits n'est pas admise. Même chose sur les stocks de médicaments. On peut discuter de l'ampleur de la mesure à prendre, mais on ne peut pas s'abriter derrière le droit européen sur cette question, car ce que nous avons proposé est le dispositif mis en place par la Finlande. Or, que sache, bien membre de l'Union européenne, et elle n'est pas en conflit avec Bruxelles sur son dispositif. Ne vous abritez pas derrière l'Union européenne pour refuser une mesure essentielle à la sécurité sanitaire de nos concitoyens qui vivent les pénuries de médicaments. Sur la question des TO-DE, je souscris aussi à ce qui a été dit dans cet hémicycle. Vous avez jugé que c'était trop coûteux pour les finances sociales, mais, en même temps, vous les dégradez volontairement. Vous le savez bien, le dispositif, de toute façon, perdurera. Je ne m'étendrai pas sur l'ensemble des questions, notamment sur le fait que tous les progrès relatifs aux outre-mer ou aux sapeurs-pompiers ont été également écartés. À l'arrivée, ce budget reste un budget d'injustice sociale. Nous ne voterons pas la question préalable, car nous sommes prêts à continuer à débattre de ce texte, mais je dois dire que les arguments en faveur de cette question sont signifiants. La parole

La crise liée à l'épidémie de covid-19 a bouleversé l'économie de notre pays, particulièrement ses finances sociales. Le Gouvernement a dû réviser trois fois les tableaux d'équilibre de 2020 et 2021, à savoir en première lecture à l'Assemblée nationale, puis, au Sénat, et, enfin, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, pour tenir compte des effets du nouveau confinement. En responsabilité, le groupe Les Républicains a adopté ces tableaux d'équilibre présentant des déficits historiques. Nous avons, en effet, considéré que l'urgence était de tout faire pour répondre par la solidarité nationale à ceux que la crise privait de leur emploi ou de revenu. Ainsi, des dispositions, modifiées au Sénat, facilitent l'accès au dispositif d'exonération en retenant un seuil unique de perte de chiffre d'affaires, qui doit être au moins égale à 50 %, pour l'ensemble des entreprises relevant des secteurs dits S1 et S1 , comme cela avait été proposé par la commission des affaires sociales. Par ailleurs, nous constatons que l'Assemblée nationale a rejoint le Sénat, et c'est tant mieux, sur l'urgence d'accélérer les réflexions sur la question du financement de la cinquième branche. Le principe d'une conférence des financeurs du soutien à l'autonomie chargée de formuler des recommandations sur le financement des mesures nouvelles est conservé, même si cette concertation sera opérée sous l'égide de la CNSA. Nous aurons donc des éléments précis d'ici au 1 mars 2021 sur les moyens nouveaux qui pourront être affectés à cette branche. Après ces notes positives, permettez-moi d'exprimer notre regret quant à la suppression de nombreuses propositions portées par nos collègues ou par la commission des affaires sociales. Nous regrettons ainsi la suppression de plusieurs mesures qui nous paraissaient opportunes, comme : la pérennisation du dispositif d'exonération TO-DE, que mes collègues ont déjà évoqué la baisse des charges sociales pour les médecins exerçant dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ; la création d'un statut de junior-entrepreneur ; ou les dispositifs relatifs à la fixation des prix des médicaments. Nous regrettons également la suppression de la mesure structurelle dont l'objectif était d'acter la nécessité de redresser les comptes du système de retraite. Depuis plusieurs années, la majorité sénatoriale plaide pour un relèvement progressif de l'âge minimum légal de la retraite, seul à même de rétablir une trajectoire financière positive pour la branche vieillesse. Cette année, nous avons proposé un dispositif très progressif, prévoyant notamment la réunion d'une conférence de financement chargée de formuler des propositions autour des différents paramètres de calcul des pensions. Selon les dernières estimations du Conseil d'orientation des retraites, la fin du déficit s'éloigne encore pour notre système des retraites. Il ne devrait pas revenir à l'équilibre avant le milieu des années 2030, dans l'hypothèse la plus favorable. Est-ce vouloir punir nos concitoyens que de constater que, par rapport au début des années 1980, l'espérance de vie des Français a progressé de sept années, alors que leur âge de départ à la retraite est avancé de trois ans, voire de quatre ou cinq ans pour ceux qui bénéficient d'un départ anticipé ? C'est pourquoi il nous semble que, sur l'exemple des régimes complémentaires, avec souplesse et pragmatisme, il faudra adapter les paramètres qui régissent aujourd'hui les conditions de départ à la retraite. Mes chers collègues, si des mesures paramétriques ne sont pas prises dans un avenir proche, les retraités d'aujourd'hui verront leur pension baisser et les futurs retraités auront des retraites beaucoup plus faibles. La paupérisation des retraités, nous n'en voulons pas ! Nous pensons que les Français sont prêts à entendre un discours de vérité. Concernant la branche maladie, les constats ne sont pas plus encourageants : le déficit de 33,7 milliards d'euros est historique ; le prévisionnel pour 2021, estimé à 23,7 milliards, ne nous invitent pas à l'optimisme. Ce déficit record est bien sûr en partie lié à la pandémie et aux conséquences budgétaires du Ségur de la santé, Ségur de la santé, auquel les professions libérales ont eu le sentiment de ne pas être assez associées. À ce titre, les médecins libéraux ont formulé le constat d'un PLFSS centré sur la crise de l'hôpital et non sur la médecine de ville. Afin de répondre en partie au mécontentement de ces acteurs essentiels du monde de la santé, qui sont, je le regrette, parfois sortis du radar du ministère, le Sénat avait voté l'avancement de la convention médicale à mars 2022, au lieu de mars 2023, comme prévu initialement dans le texte. Malheureusement, vous n'avez pas jugé pertinent de trouver une solution de compromis et ainsi d'apaiser les légitimes inquiétudes formulées ces derniers mois. Le domaine hospitalier n'est pas en reste, puisque ce texte contient deux mesures qui vont à l'encontre de l'esprit initial de l'assurance maladie premièrement, le financement du volet hospitalier du plan de relance par l'assurance maladie, alors que cela devrait relever de la mission « Plan de relance » dédiée au sein du budget général ; deuxièmement, et c'est un sujet qui fâche, la reprise de la dette des établissements de santé assurant le service public hospitalier, qui devrait non pas alourdir les déficits sociaux, mais plutôt se faire par le biais de crédits budgétaires. J'attire particulièrement votre attention sur ce dernier point, qui est, en partie, la cause de En effet, nous étions prêts à faire de nombreuses concessions si des garanties avaient été présentées concernant la reprise de la dette hospitalière. Je le répète une nouvelle fois : l'assurance maladie, via la Cades, n'a pas vocation à se substituer à l'État concernant la gestion financière des hôpitaux. Ce n'était pas le cas en 1945 lors de la création de l'assurance maladie

Vous l'aurez compris, madame la ministre, ce PLFSS 2021 nous laisse un sentiment de rendez-vous manqué avec les acteurs de la santé et avec la santé des acteurs du quotidien. Nous regrettons l'absence de cap, de vision, de cohérence dans l'ensemble de ces mesures.

Parfois généreux avec le secondaire, souvent avares avec l'essentiel, vous avez manqué de recul face à une situation inédite et dramatique, qui laissera des traces indélébiles dans notre société et sur notre économie. Certaines mesures votées dans le cadre de ce texte doivent nous interroger sur la définition même d'une loi de financement de la sécurité sociale. Vous auriez pu vous appuyer sur la sagesse du Sénat, mais vous ne l'avez pas fait. Vous auriez pu être ambitieux sur de nombreuses mesures, en rappelant aux Français que ces avancées ont un coût important et qu'elles nécessitent une contrepartie de leur part, mais vous ne l'avez pas fait. Vous préférez vous satisfaire de quelques totems obtenus aux dépens des générations futures, qui devront payer une addition plutôt salée. Nous comprenons la gravité de la situation actuelle et des choix cornéliens que vous avez dû faire ces derniers mois, et que vous continuerez à faire tant que cette pandémie ne sera pas endiguée. À cet égard, le Sénat a toujours fait le choix de la modération et du dialogue. Nous vous avons donné les moyens de lutter contre les effets de la pandémie. C'est pourquoi, dans un souci d'intérêt général, je vous demande, pour l'avenir, d'être plus attentifs à la voix du Sénat, qui, je le sais, apporte sagesse et hauteur de vue dans le débat public. Cependant, pour toutes les raisons évoquées précédemment, et parce que la reprise de la dette hospitalière par la Cades est un point non négociable, le groupe Les Républicains votera la motion tendant à opposer la question préalable proposée par la commission des affaires sociales. La parole

prononcés le 16 juillet dernier devant le Sénat : « Si j'ai tenu à présenter la politique de mon gouvernement devant le Sénat, c'est avant tout pour marquer mon attachement personnel, peut-être familial aussi, au bicamérisme et à l'équilibre démocratique qu'il garantit. Devant vous, comme hier

en avons discuté en commission des affaires sociales, cette bonne volonté n'était pas réciproque. Ce n'est pas forcément nouveau dans la V République, mais ce n'est pas une raison pour s'en satisfaire.

nous avions adoptés sur l'initiative de notre groupe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même ! Je serai quelque peu didactique et citerai certains de nos collègues. Je pense d'abord aux services à la personne. Notre collègue Françoise Gatel avait fait adopter deux amendements dans ce domaine. Le premier, objet la notion de « domicile à usage privatif », qui n'est pas définie en droit de la sécurité sociale, ce qui a amené certaines Urssaf à rejeter les demandes d'exonération de certaines catégories d'établissements, au motif qu'il ne s'agirait pas « strictement » d'un domicile privatif. Cette disposition n'a pas

J'avais fait adopter, avec mes collègues, une disposition permettant de soutenir ce secteur. Sans remettre en cause le principe de régulation de ce secteur, nous constations que les dispositifs médicaux se voient appliquer une clause de sauvegarde inadaptée aux spécificités du secteur.

encore aux maisons de naissance et aux sages-femmes. Notre collègue Élisabeth Doineau avait fait adopter deux amendements relatifs aux maisons de naissance. Le premier visait à renforcer l'autonomie des sages-femmes dans les domaines médicaux, administratifs et financiers lorsqu'elles exercent dans une maison de naissance ; le second, à comptabiliser l'activité des maisons de naissance avec celle de leur structure partenaire. Concernant les services d'urgence, notre collègue Michel Canevet avait fait adopter un amendement visant à mettre en oeuvre une expérimentation permettant d'améliorer la régulation des patients au sein de ces services, un nombre important de passages pouvant être redirigés vers la médecine

pour cause de maternité ou de paternité. Cet avantage ne bénéficie actuellement qu'aux médecins conventionnés. Madame la ministre, mes chers collègues, vous comprendrez le regret

Les principaux articles de ce texte, les tableaux d'équilibre, la trajectoire pluriannuelle et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ont été rectifiés à plusieurs reprises, dans chacune des chambres en première lecture, puis de nouveau à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Ce texte est inédit par l'ampleur des déficits et l'incertitude qui s'attache à leur évolution. Ces déficits abyssaux et la probabilité qu'ils se creusent encore davantage, le Sénat les a acceptés. Il a soutenu les efforts déployés par le Gouvernement pour tenter d'éviter que notre économie, mise à mal par les restrictions liées à la crise sanitaire, ne sombre. Ces efforts se traduisent par une plongée vertigineuse des finances publiques, qui n'étaient qu'à peine convalescentes. Devant ce constat, le Sénat a porté deux messages principaux. exprime la nécessité de réaffirmer et de préserver, le moment venu, l'objectif du redressement de la trajectoire de nos comptes sociaux. Il tient à une raison très simple : les dépenses sociales sont des dépenses de transfert ; si elles dérapent durablement, c'est le système tout entier qui risque l'effondrement. Tel n'est pas notre choix : nous tenons à un modèle social solidaire. Pour le préserver, il faut le financer. Ce premier message s'est traduit par l'adoption d'un amendement au rapport figurant en annexe B, qui décrit la trajectoire pour les cinq années à venir sans porter aucune trace de redressement après 2022. Il s'est également traduit par l'adoption d'un amendement portant sur la question des retraites. Notre système de retraites a fait l'objet de nombreuses réformes dites « paramétriques ». Ce qualificatif n'est en rien péjoratif, s'agissant d'un risque qui se pilote bien par trois paramètres : le niveau des cotisations, celui des pensions et la durée pendant laquelle elles sont servies. Avant que la crise sanitaire n'interrompe le processus, le Sénat devait bien examiner un projet de réforme des retraites, prévue à l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. Une conférence des financeurs devait examiner les moyens de parvenir à l'équilibre à l'horizon de 2025 pour l'entrée en vigueur de la réforme systémique, en agissant sans doute sur certains paramètres. Le Sénat a voulu relancer ce processus, car nous savons que la réforme est nécessaire, qu'elle le sera plus que jamais demain et qu'elle sera d'autant plus douloureuse qu'elle aura trop tardé. Pour autant- cela m'amène au second message porté par notre institution -, s'il faut impérativement réformer, il faut le faire dans un cadre clair et pour de bonnes raisons. En d'autres termes, s'il faut demain réformer les retraites, ce n'est pas parce que l'assurance maladie a dû payer les masques de Santé publique France. S'il faut augmenter la contribution au remboursement de la dette sociale, ce n'est pas parce que la Cades se finance sur les marchés pour permettre aux hôpitaux d'investir. C'est pour ces raisons que le Sénat a refusé les modalités de reprise d'une partie de la dette des hôpitaux. Ce ne sont pas des raisons théoriques : elles ont une portée pratique et très politique. Nous sommes finalement favorables à la règle du « chacun chez soi », mantra du précédent Gouvernement pour justifier une ponction sur des excédents de la sécurité sociale qui ne se sont malheureusement jamais matérialisés. Elle suppose de revenir aux fondamentaux des assurances sociales, en clarifiant les financements en fonction des risques couverts accidents du travail, chômage et retraites se financent par des cotisations qui ont une contrepartie en prestations. C'est le sens de la loi Veil de 1994 : les allégements sans compensations ne produisent que des déficits. En dépit des critiques adressées au pilotage de la sécurité sociale, celui-ci n'a pas perdu de vue l'objectif de l'équilibre, à la différence du budget de l'État. Nous ne devons pas le perdre de vue non plus ; nous pensons qu'il serait illusoire, voire dangereux, de prétendre pouvoir à terme nous en dispenser. Ayant constaté un désaccord sur tous ces points avec le Gouvernement et l'Assemblée nationale, la commission des affaires sociales a considéré avoir épuisé le dialogue institutionnel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

de la majorité présidentielle pour le débat démocratique et le travail parlementaire, mépris que l'examen de ce texte à marche forcée illustre tant sur le fond qu'à travers la méthode.

a ainsi trahi un flagrant dédain envers ce qui ne vient pas d'elle. Il s'agit d'un jusqu'au-boutisme aveugle, alors même que, depuis le début des crises que traverse notre pays, le Président de la République multiplie les appels à l'unité nationale. En même temps, votre majorité bafoue le rôle du Parlement

Évidemment, pour celles et ceux qui considèrent le Parlement comme une simple chambre d'enregistrement, il n'y a là rien de surprenant ! Autant vous dire que telle n'est pas notre conception du travail parlementaire. Vous l'aurez compris : ulcérés par un fond dogmatique et par les procédés péremptoires de l'exécutif et de sa majorité, les sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'abstiendront sur cette motion, pour les raisons

Je regrette qu'aujourd'hui le Sénat ne veuille pas débattre et montre aux Français le peu d'intérêt du débat démocratique. On a le droit de rigoler ? La parole est à Mme Véronique

Le scrutin est ouvert.

rejeté. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires européennes a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.